La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

a caricaturé un vote unanime du Sénat hier après-midi. Cette déclaration me paraît en contradiction avec les propos tenus par le Président de la République et le Premier ministre, qui disaient avoir entendu et compris ce sentiment d'abandon et de lassitude qui gagne les maires, en particulier ceux des petites communes, mais pas qu'eux. Pour retrouver la sérénité de nos débats, j'ai donc souhaité savoir si la position exprimée par le ministre de l'action et des comptes publics reflétait l'état d'esprit du Gouvernement vis-à-vis des élus locaux, qui, vous le savez, font preuve de dévouement au service de nos concitoyens. Sur son appel, je me suis entretenu hier soir avec le Premier ministre, qui m'a fait part de sa volonté d'apaisement, avec les élus locaux comme avec la représentation nationale. Le Gouvernement, par la voix du ministre chargé des relations avec le Parlement, que je remercie, a confirmé qu'il ne s'agissait pas de sa position, confirmant du même coup ce que m'avait dit le Premier ministre, et a rappelé qu'il était attentif aux travaux du Sénat sur la question du statut, dont la revalorisation du mandat. « La France ne serait pas la même sans ses maires. [ ...] Être aux côtés des maires de France, c'est être aux côtés des Français », écrivait le Président de la République dans sa lettre à tous les maires de France, le 16 novembre dernier. Si l'on veut pouvoir restaurer un dialogue sain et serein entre les élus locaux, les élus territoriaux et l'État, il faut commencer par témoigner du respect, passer aux actes et respecter la représentation nationale. Ce tweet est une ministérielle,

jusqu'à ce que le Gouvernement ait informé le Sénat du retrait de ce tweet. Alors, nos travaux pourraient se poursuivre. Je porterai une attention toute particulière à un principe pour moi essentiel au Sénat, que je rappelle à chacune